prises pour son application, la commission de l'aménagement du territoire a émis, lors de sa réunion du 9 juillet 2019, un avis favorable- 14 voix pour, 1 voix contre -à la nomination de M. Laurent Hénart aux fonctions de président du conseil d'administration de Voies navigables de France. Par ailleurs, conformément aux mêmes dispositions, elle a émis un avis favorable- 18 voix pour -à la reconduction de Mme Catherine Guillouard aux fonctions aux fonctions de président-directeur général de la Régie autonome des transports parisiens. L'ordre du jour appelle la discussion, en nouvelle lecture,

Madame la présidente, madame la présidente de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, chère Catherine Morin-Desailly, monsieur le président de la commission de la commission des finances, monsieur le président de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, cher Jean-Pierre Leleux, monsieur le rapporteur de la commission de la culture, de l'éducation et de la communication, cher Alain Schmitz,

de la cathédrale Notre-Dame de Paris, voilà bientôt deux mois, notre objectif n'a pas changé. Il s'agit d'offrir à Notre-Dame une restauration à sa hauteur, à la hauteur de ce qu'elle représente et de ce qu'elle symbolise, pour notre pays et son patrimoine ou, plus largement, pour le monde entier. Dès le soir du 15 avril, une mobilisation sans précédent s'est enclenchée. Une fois encore, je veux remercier toutes celles et tous ceux qui y ont participé les sapeurs-pompiers de Paris, aidés et renforcés par leurs collègues des autres départements d'Île-de-France ; les policiers ; les gendarmes ; les agents du ministère de la culture ; ceux de la Ville de Paris et du diocèse ; mais aussi les experts, les institutions et entreprises qui ont donné ou promis de donner et proposé d'aider à la restauration. J'y ajoute, évidemment, les centaines de milliers de particuliers qui, en France et de par le monde, ont souhaité donner dès le soir de l'incendie. Ainsi les dons ont-ils afflué, rapidement et en nombre.

C'est tout le sens du projet de loi qui vous est présenté. Ce texte nous permet d'encadrer la souscription nationale annoncée par le Président de la République : tant le mécanisme de collecte que le dispositif fiscal afférent, ainsi que leurs modalités de suivi et de contrôle. Depuis votre première lecture de ce texte, il me semblait important de revenir à son esprit initial. L'objet de la loi, en effet, n'est pas de préempter un débat patrimonial. Je trouve sain que ce débat ait lieu. Je trouve sain qu'on parle avec ferveur de patrimoine et de culture. Je trouve sain que les Français se sentent si concernés par les monuments que l'histoire leur a légués.

amorcée ; nous sommes toujours dans la phase de consolidation et de conservation. La semaine dernière, des cintres ont été installés- peut-être avez-vous assisté à cette scène assez spectaculaire -pour soutenir les arcs-boutants de la cathédrale,

Non, l'objet du projet de loi, c'est d'abord et avant tout la souscription nationale. Le texte qui vous est présenté aujourd'hui le réaffirme clairement. Je vous le disais en première lecture : nous voulons aller vite, mais sans, pour autant, nous précipiter. L'objectif fixé par le Président de la République de restaurer Notre-Dame de Paris en cinq ans est ambitieux et volontariste. Il permet de motiver les équipes et mobiliser l'ensemble des acteurs concernés. Mais je le réaffirme ici : jamais, dans cette restauration, nous ne confondrons vitesse et précipitation. Néanmoins, la situation de Notre-Dame nous imposait deux temporalités. D'une part, il y avait urgence- il y a toujours urgence -à organiser le dispositif de la souscription nationale et ses modalités ; d'autre part, s'agissant de l'organisation du chantier de restauration, il fallait prendre le temps de la réflexion pour travailler avec l'ensemble des ministères concernés, pour identifier, ensemble, les assouplissements et adaptations à prévoir et pour définir l'organisation optimale permettant de mener à bien ce chantier au regard des objectifs fixés. Lors de la première lecture, je vous avais indiqué que le Gouvernement s'attelait à définir au plus vite cette organisation. Je m'y étais engagé, et je suis heureux de me présenter de nouveau devant vous, car, depuis lors, nous avons énormément Suffisamment, en tout cas, pour remplacer l'habilitation à légiférer par ordonnance initialement prévue à l'article 8 par une inscription dans la loi elle-même du statut de l'établissement public, ce qui permet de soumettre ce texte à votre examen. Suffisamment, aussi, pour inscrire dans la loi une partie importante des adaptations du droit rendues nécessaires par le chantier exceptionnel, adaptations prévues à l'article 9. Je reviendrai sur ces deux points. avant de vous en exposer les grandes lignes, il me semble important de réaffirmer les principes essentiels du projet de loi, qu'il importe de préserver. Ce texte nous permet, à la fois, d'encadrer la souscription nationale dédiée, en fixant par la loi les règles qui lui sont applicables, et d'apporter des garanties de sécurité et de transparence aux centaines de milliers de donateurs, Français ou étrangers. Cette transparence, nous la leur devons. Les donateurs ne seront pas trahis : leurs dons iront bien à Notre-Dame de Paris. Nous y veillerons ; soyez-en assurés

pour ne pas dire exagéré, de parler de « sur-collecte » dans le cadre de la souscription. En outre, le coût total des travaux n'a pas encore été chiffré. Pour l'instant, les travaux portent seulement, comme je l'ai indiqué au début de mon propos, sur la mise en sécurité de l'édifice.

Pour opérer cette souscription nationale, outre les versements directs à l'État, nous avons pu compter depuis le 16 avril sur la mobilisation de trois fondations reconnues d'utilité publique- la Fondation de France, la Fondation du patrimoine et la Fondation Notre-Dame que sur celle du Centre des monuments nationaux, opérateur bien connu du ministère de la culture. Je veux sincèrement les en remercier.

sera mis en place, réunissant le Premier président de la Cour des comptes et les présidents des commissions chargées des finances et de la culture du Sénat et de l'Assemblée nationale, ou leurs représentants.

Par ailleurs, l'examen en première lecture nous a permis de renforcer la transparence quant au suivi de la souscription et de l'application du dispositif fiscal afférent. C'est une transparence à l'égard du Parlement, tout d'abord. L'article 5 dispose ainsi que le Gouvernement lui rendra compte, dans un rapport, de la part et du montant des dons effectués au titre de la souscription nationale ayant donné lieu à une réduction d'impôt, et de la participation des collectivités territoriales. C'est une transparence à l'égard du public, aussi. L'article 7 impose désormais la publication d'un rapport sur la collecte des fonds, leur provenance et leur affectation. Concernant l'affectation des fonds, justement, je tiens à rappeler que le projet de loi dont nous allons débattre ne portera évidemment pas atteinte aux principes des lois de 1905 et de 1907 : ni au principe de laïcité ni aux droits du culte affectataire, c'est-à-dire à la répartition des prérogatives et responsabilités entre l'État et le diocèse de Paris. L'intégralité des dons en faveur de la restauration de Notre-Dame de Paris passera ainsi par la souscription nationale, à l'exception de ceux qui ont spécifiquement pour objet de financer la restauration des biens appartenant au diocèse ou, plus généralement, les besoins relevant de l'exercice du culte. Ce projet de loi, je le disais, doit garantir la transparence de la souscription nationale.

Dans la limite de 1 000 euros, le taux de réduction d'impôt sur le revenu au titre des dons et versements effectués par les particuliers en faveur du trésor public, du Centre des monuments nationaux et des trois fondations reconnues d'utilité publique est porté de

Les collectivités territoriales et leurs groupements pourront aussi participer au financement des travaux, au-delà de leur périmètre de compétence territoriale. L'article 4 lève toute incertitude éventuelle tenant aux règles habituelles de compétence ou à la condition d'intérêt local. Les dépenses des collectivités en faveur de Notre-Dame seront considérées comme des dépenses d'équipement. Elles ne seront donc pas prises en compte pour appréhender le plafond annuel d'évolution des dépenses de fonctionnement de 1,2 %. Voilà pour ce qui concerne la souscription nationale, dont les grandes lignes n'ont pas changé depuis l'examen en première lecture du texte. Pour autant, depuis lors, comme je m'y étais engagé, le Gouvernement a poursuivi ses travaux pour préciser le projet de loi. de loi. Il a défini l'organisation pour mener à bien les opérations de restauration et de conservation. En vertu de l'article 8, un établissement public de l'État à caractère administratif sera créé. Sa mission première sera d'assurer la maîtrise d'ouvrage. Les fonds issus de la souscription nationale serviront aussi à financer son fonctionnement. Il sera placé sous la tutelle du ministère de la culture- c'est vous, mesdames, messieurs les sénateurs, qui avez apporté cette précision au texte et je tiens à le saluer. Comme l'a annoncé le Président de la République, voilà quelques semaines, à l'occasion de la remise du prix Pritzker, l'établissement public sera également en charge de réaliser les travaux d'aménagement de l'environnement immédiat de la cathédrale, à savoir, principalement, le parvis, le square Jean-XXIII, la promenade du flanc sud de l'île de la Cité. Toutefois, nous ne trahirons pas les donateurs si la compétence de l'établissement public est étendue à l'environnement immédiat de Notre-Dame, la souscription nationale, elle, ne concerne que la cathédrale, sans inclure l'aménagement de cet environnement. La Ville de Paris et le culte affectataire seront associés à la gouvernance de l'établissement public, de par la composition de son conseil d'administration. La situation des riverains et des commerçants sera prise en compte. C'est encore vous, mesdames, messieurs les sénateurs, qui avez apporté cette précision au texte, et je vous en remercie. L'avis des professionnels du patrimoine sera également pris en compte. C'est tout le sens du conseil scientifique de l'établissement public. Consulté régulièrement, il sera le garant de la qualité scientifique et historique de la restauration. En parallèle, la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture, la CNPA, sera évidemment consultée sur l'avancée des travaux et les choix de restauration.

Je tiens à remercier ses membres de leurs travaux fructueux, de leur vigilance et de leur attention sans cesse renouvelée à notre patrimoine et, en l'occurrence, à la cathédrale. Nous avons par ailleurs précisé, à l'article 9, les assouplissements aux législations en vigueur. Ces assouplissements, je m'y étais engagé, seront strictement proportionnés aux besoins du chantier. Il n'est pas question de se servir de la restauration de Notre-Dame pour piétiner, de quelque manière que ce soit, le droit français et européen du patrimoine, de l'environnement, ou de l'urbanisme. Cela n'a jamais été l'intention du Gouvernement. En tant que ministre de la culture, je serai le garant inlassable de l'occasion de le dire en première lecture. Nous avons de ce fait inscrit dans la loi les dérogations en matière de patrimoine. Elles permettront de confier à l'Institut national de recherches archéologiques préventives, l'Inrap, la réalisation des fouilles archéologiques rendues nécessaires dans le cadre des travaux. des travaux. Elles permettront de réduire la durée d'instruction des autorisations d'installation temporaire, en supprimant la consultation de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, la CRPA, en cas de recours contre la position de l'architecte des bâtiments de France.

commercial. Seuls les dispositifs visant exclusivement à informer le public sur les travaux seront autorisés. Vous aviez exprimé vos craintes sur ce sujet en commission ; nous les avons entendues. Nous avons également veillé à circonscrire le champ des dérogations nécessaires par ordonnance, concernant les questions de voirie, d'urbanisme et d'environnement. Sur ces sujets, établir les dérogations demande effectivement une connaissance précise du projet de restauration,

Madame la présidente, monsieur le ministre, madame la présidente de la commission, mes chers collègues, en première lecture, le Sénat avait déploré la précipitation avec laquelle le projet de loi avait été élaboré et regretté qu'il s'apparente, à plusieurs égards, à une loi d'exception. Le travail minutieux que nous avions alors réalisé avait permis de modifier le texte, afin de garantir l'exemplarité du chantier de Notre-Dame, compte tenu de son caractère emblématique, et de sécuriser le cadre légal offert aux donateurs, de manière à leur apporter des garanties suffisantes pour permettre à l'élan de générosité de se poursuivre. Malheureusement, l'inflexibilité dont vous avez fait preuve en première lecture, monsieur le ministre, comme l'intransigeance de la majorité présidentielle au moment de la commission mixte paritaire, ne nous a pas permis d'aboutir à l'élaboration d'un texte commun. Notre volonté de supprimer l'article 9, pourtant justifiée par les risques que ce dernier faisait courir sur la crédibilité de notre législation et le précédent qu'il risquait de constituer à l'avenir, n'a pas fait l'objet d'un consensus parmi les députés. Que penser du texte résultant des travaux de l'Assemblée nationale ? La réponse n'est pas évidente, car les discussions en nouvelle lecture ont connu un véritable tournant en séance publique. Sans surprise, la commission des affaires culturelles de l'Assemblée nationale a, dans un premier temps, rétabli l'essentiel du texte qu'elle avait adopté en première lecture, balayant les dispositions introduites par le Sénat tendant à enrichir, à préciser et à sécuriser juridiquement les articles du projet de loi. Tout au plus a-t-elle adopté sans modification l'article 8 , que nous avions introduit en séance publique sur l'initiative de notre collègue Jean-Pierre Leleux, pour garantir l'information et la consultation de la Commission nationale du patrimoine et de l'architecture sur l'avancement des études et des travaux du chantier de Notre-Dame. C'est une bonne chose, puisque cet article, qui n'a pas davantage été amendé en séance publique, est désormais conforme et fera partie de la loi promulguée. En revanche, si je me fie à mes collègues bien plus expérimentés que moi dans l'univers parlementaire, l'inflexion qu'a connue le texte en séance publique est absolument inédite, après le refus de compromis auquel nous nous étions heurtés lors des précédentes phases de la procédure législative. Contre toute attente, en effet, le Gouvernement a effectivement déposé deux amendements visant à complètement remanier la rédaction des articles 8 et 9 du projet de loi. Quel revirement inattendu sur deux articles qui figuraient parmi les plus sensibles ! Même si nous ne pouvons que regretter l'intervention de ces modifications à un stade aussi avancé de la procédure législative, il nous faut reconnaître qu'elles rejoignent plusieurs des préoccupations exprimées par le Sénat. La nouvelle rédaction de l'article 8 met fin à l'ambiguïté que nous avions dénoncée en première lecture, puisque celui-ci confie définitivement à un nouvel établissement public, à caractère administratif et placé sous la tutelle du ministère de la culture, comme nous le demandions, le soin d'assurer la maîtrise d'ouvrage des travaux de restauration de Notre-Dame.

ainsi qu'à l'identification des besoins de formation professionnelle pour les travaux de restauration de l'édifice et à la médiation et valorisation du chantier, ce que le Sénat avait soutenu en première lecture. demandé à l'établissement public de prendre en compte la situation des commerçants et des riverains, comme y avaient appelé les élus parisiens. La nouvelle rédaction de l'article 9 restreint considérablement le champ de l'habilitation à déroger aux règles de droit commun par ordonnances pour faciliter l'exécution du chantier de Notre-Dame. Comme nous l'espérions, les dérogations au code du patrimoine, au code général de la propriété des personnes publiques et aux règles de publicité prévues par le code de l'environnement sont désormais listées à l'article 9 et ne font plus l'objet d'une habilitation. En revanche, une habilitation demeure pour permettre au Gouvernement de déroger par ordonnances aux règles en matière de voirie, d'environnement et d'urbanisme, et d'adapter les règles applicables aux travaux et aux opérations connexes pour faciliter la construction de bâtiments nécessaires au chantier, ainsi que son approvisionnement et l'accueil du public. Que penser de ces évolutions ? Je crois que nous pouvons légitimement y voir la preuve du bien-fondé des propositions que nous avions formulées en première lecture et peut-être, aussi, un aveu d'une certaine précipitation dans l'élaboration du texte. Doit-on s'en satisfaire ? Je ne vous surprendrai pas, monsieur le ministre, en vous disant que la réponse à cette question est en demi-teinte. Oui, ces évolutions améliorent le texte par rapport à la version qui nous avait été soumise en première lecture. Mais elles restent, à nos yeux, nettement insuffisantes. À l'article 8, compte tenu de la mission confiée à l'établissement public, à savoir « assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations concourant à la conservation et à la restauration de la cathédrale des doutes importants subsistent sur la répartition des compétences entre maîtrise d'ouvrage et maîtrise d'oeuvre. Le texte ne sera pas clair, à nos yeux, tant qu'il ne précisera pas que la maîtrise d'oeuvre restera exercée sous l'autorité de l'architecte en chef des monuments historiques. Il nous paraît également important d'encadrer la durée du fonctionnement de l'établissement public. Rien ne justifie qu'il perdure une fois les travaux liés au sinistre et à l'aménagement des abords immédiats de la cathédrale achevés. À l'article 9, nous jugeons dangereux de dispenser le préfet de région de consulter la CRPA avant de rendre sa décision concernant un recours formé par l'autorité compétente pour les autorisations de travaux contre l'avis d'un Outre le signal négatif que cette dérogation constituerait en matière de protection du patrimoine, il y a en l'espèce un vrai risque de faire perdre tout son sens à la procédure de recours, en abandonnant la consultation de la CRPA, puisque la même autorité, à savoir le préfet, est à la fois chargée de délivrer les autorisations de travaux liés à la conservation et à la restauration de la cathédrale et de statuer dans le cadre du recours. Compte tenu de l'opposition que nous avions manifestée en première lecture à la perspective d'une loi d'exception, le maintien d'une habilitation au Gouvernement à légiférer par ordonnances pour déroger aux règles de droit commun, quand bien même ce serait sur un champ plus réduit qu'en première lecture, nous paraît toujours inacceptable. Nous regrettons que vous n'ayez toujours pas clairement motivé ces dispositions, et j'espère que nos débats de ce jour pourront enfin nous apporter quelques éclairages. Sur tous les autres articles du projet de loi, l'Assemblée nationale est revenue presque intégralement au texte qu'elle avait adopté en première lecture. C'est ce qui a justifié notre décision de rétablir en commission plusieurs des dispositions adoptées par nos soins en première lecture. Ces dispositions nous paraissent indispensables pour garantir l'équilibre et la sécurité juridique du projet

plutôt que d'inscrire expressément cette date dans la loi ? Reconnaissez tout de même que cela simplifierait grandement les choses et permettrait que les pratiques que vous entendez mettre en oeuvre soient conformes au droit que nous sommes en train d'élaborer.

l'on constate que le bien « Paris, rives de la Seine » n'est toujours pas doté d'un plan de gestion, alors que cette obligation figure dans la loi depuis trois ans déjà et émane des mêmes recommandations de l'Unesco, on est enclin à penser qu'il n'est pas inutile d'insister sur cette question. La restauration de Notre-Dame n'est pas un chantier anodin. Nous savons tous combien notre pays va être observé à cette occasion, sachant que les donateurs étrangers- vous l'avez rappelé, monsieur le ministre -se sont fortement mobilisés. Nous sommes fiers que l'expertise de la France en matière de protection du patrimoine soit ainsi reconnue de par le monde. C'est pourquoi nous sommes convaincus que cette restauration doit être opérée dans le cadre des règles internationales et nationales en vigueur.

Vous nous avez dit à plusieurs reprises que leurs versements dans le cadre de la souscription seront considérés comme des subventions d'investissement. Dès lors, comment interpréter le fait que vous demandiez une nouvelle fois la suppression de cette disposition que nous avons rétablie ? Cette attitude ne nous semble pas de bon aloi, si votre souhait est de sécuriser les dons des collectivités territoriales, qui, pour beaucoup, sont revenues ou reviennent sur leurs promesses. Monsieur le ministre, j'espère que le présent débat nous permettra de rétablir un dialogue fécond sur ce texte et que la voix du Sénat, qui a enfin commencé à porter la semaine dernière à l'Assemblée nationale, continuera de vous convaincre, afin de conforter l'exemplarité du chantier de Notre-Dame et de notre régime juridique de protection du patrimoine. Ces derniers, me semble-t-il, auraient davantage mérité de faire l'objet d'un consensus depuis le début de nos discussions

avons reçues, cette précipitation contraste avec le manque d'empressement de l'État à régler les factures des entreprises qui interviennent sur Notre-Dame depuis le sinistre. Prenons garde à ne pas mettre en danger les savoir-faire dont nous allons avoir besoin dans les mois et années à venir et que nous voulons voir valorisés à l'occasion du chantier. ! En découvrant le présent texte, nous avions tenu à le dire : très peu de ces dispositions justifient le recours à une loi. Une souscription nationale aurait très bien pu être ouverte par décret. Les services du ministère de la culture ou certains des établissements placés sous sa tutelle auraient pu prendre en charge la maîtrise d'ouvrage des travaux. Quant à notre législation actuelle, elle ne s'est jamais révélée un obstacle pour mener à son terme un chantier de restauration : les collectivités territoriales, que nous représentons, pourraient en témoigner.

dont l'utilité n'est pas avérée, et qui, dans le même temps, crée une Agence nationale du sport sans se rendre compte qu'il aurait fallu passer par la loi pour déterminer les modalités de son fonctionnement ... Très bien ! De mémoire de sénatrice, je n'avais jamais connu autant de bizarreries et d'incohérences dans la procédure législative. depuis le début de l'examen de ce texte, nous nous sommes heurtés à des refus catégoriques de prise en compte de notre travail, pourtant minutieux et équilibré.

les députés de la majorité ont refusé de prolonger les débats au-delà de la discussion générale, sans guère d'explications quant aux raisons de leur intransigeance. Pourtant, le patrimoine est habituellement un sujet de consensus. Dans ce contexte, nous n'avons pas été surpris de constater que nos collègues députés avaient décidé, en nouvelle lecture, de rétablir leur texte de première lecture presque à l'identique.

Ces inflexions vont dans le sens de la préservation de notre État de droit, sur laquelle nous n'avons cessé d'alerter. Dès lors, pourquoi ne pas nous suivre davantage, aller au bout de notre logique pour garantir un texte véritablement cohérent, rassurant et protecteur ? Pourquoi laisser planer de telles ambiguïtés dans le texte ? Pourquoi ne pas y inscrire clairement que l'architecte en chef des monuments historiques sera responsable de la maîtrise d'oeuvre ? Compte tenu du rôle dévolu à l'établissement public, également chargé de la maîtrise d'ouvrage, c'est une précision essentielle pour éviter tout mélange des genres. Pourquoi s'évertuer à considérer la cathédrale comme hors-sol, en refusant d'insérer toute référence à l'Unesco ? Franchement, je peine à comprendre la négligence que subit ce classement,

Paris, rives de la Seine » ne dispose toujours pas d'un plan de gestion, dont une disposition du code du patrimoine impose pourtant l'élaboration depuis maintenant trois ans. Pourquoi maintenir des habilitations à légiférer par ordonnances qui ne font que trahir l'impréparation du Gouvernement ?

le texte ? Les débats autour de ce projet de loi ont mis en lumière un certain nombre d'inquiétudes. La première inquiétude concerne le dispositif en matière de mécénat, que la commission des finances de l'Assemblée nationale menace de remettre à plat, comme la plupart des crédits d'impôt en matière culturelle. Notre commission de la culture s'est penchée, l'an passé, sur la question du mécénat dans le domaine culturel- M. Schmitz était d'ailleurs le rapporteur de ce elle a démontré à quel point le mécénat constituait une ressource importante pour le financement de la culture. Les acteurs culturels, à qui l'État demande depuis des années d'accroître leurs ressources propres, ne comprendraient pas qu'un dispositif devenu essentiel pour eux et ayant fait ses preuves soit remis en cause, même partiellement. Les conséquences en seraient terribles. Nous avons aussi constaté que la restauration du patrimoine fait partie des domaines des domaines du champ culturel qui attirent le plus de mécènes. Compte tenu de l'état de notre patrimoine, prenons garde à ne pas « couper le robinet » sans évaluation préalable.

Nous le savons également : les crédits de l'État dans ce domaine, même s'ils ont été légèrement redressés, ne retrouveront probablement pas les niveaux passés. Cet investissement est pourtant nécessaire pour assurer correctement la restauration de notre patrimoine et développer la culture de l'entretien, qui nous manque tant. Monsieur le ministre, j'espère que vous pourrez nous transmettre, avant la période budgétaire, le dernier

de la cathédrale Notre-Dame, ravagée par un incendie le 15 avril précédent, s'est soldée par un échec. Elle a buté sur le régime dérogatoire aux règles d'urbanisme mis en place à l'article 9, dont le Sénat avait acté la suppression. L'Assemblée nationale a finalement voté, en nouvelle lecture, des modifications significatives aux articles 8 et 9 du projet de loi. Ce faisant, elle a apporté, malheureusement de manière tardive, une réponse partielle aux préoccupations exprimées par le Sénat en première lecture. On peut regretter que l'Assemblée nationale ne soit pas allée plus loin, en reprenant l'ensemble des dispositions adoptées par le Sénat tendant à enrichir, à préciser et à sécuriser juridiquement les articles du projet de loi. Notre travail semblait pourtant intéressant pour compléter ce texte. D'ailleurs, monsieur le ministre, vos nouvelles propositions, que nous tenons à saluer, en sont la plus belle des illustrations. Néanmoins, il sera de notre devoir de contrôler, dans les mois à venir, la nature et le périmètre des ordonnances prises par le Gouvernement dans le cadre du chantier de ce monument emblématique de notre patrimoine national. Ce chantier devra être irréprochable à tout point de vue : dimension exceptionnelle et exemplarité ne devront pas s'exclure. L'établissement public qui mènera les travaux de restauration de la cathédrale devra également être exemplaire dans son travail et associer l'ensemble des parties prenantes, tout au long du chantier. La restauration de la cathédrale devra être à la hauteur de l'élan de soutien massif et inédit que nous avons connu ; à la hauteur de ce que symbolise ce joyau de notre patrimoine national. Évidemment, nous devons nous demander quelle restauration nous souhaitons pour Notre-Dame. Je suis certaine que cette question cruciale donnera lieu à de nombreux débats à tout niveau. Même s'il est clair qu'il faut préserver au maximum les traits généraux de l'édifice, il ne faudra pas manquer d'ambition pour ce chantier unique. Il faudra aussi veiller à ce que la restauration de Notre-Dame ne se fasse pas au détriment d'autres chantiers et d'autres monuments dans nos territoires. Nous le savons tous : les budgets des collectivités locales sont contraints et, bien souvent, ces dernières ne sont pas en mesure de préserver leur patrimoine comme elles le souhaiteraient. Parfois même, elles n'ont pas les moyens d'assurer les travaux d'urgence, pourtant indispensables à la préservation des édifices. Il ne faut pas négliger ce patrimoine, reflet de l'histoire de nos communes. Veillons à déployer les moyens de soutenir les collectivités territoriales dans leurs projets de préservation du patrimoine français

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans cet hémicycle comme partout, à Paris, en France et dans le reste de l'Europe, le même constat s'impose : pour parler de Notre-Dame de Paris, nul besoin d'être un spécialiste du patrimoine, de la conservation des bâtiments, de l'architecture ou de l'histoire religieuse de notre pays. Nul besoin non plus de se référer à des plans ou à des documents photographiques, de se plonger dans des ouvrages savants renvoyant à l'édification minutieuse de ce formidable monument. Non, il nous suffit pour une fois de fermer les yeux. Faites-en l'expérience, mes chers collègues. Fermez les yeux et vous verrez ! Instantanément, votre affect personnel imprimera sur votre rétine et dans votre esprit l'image de Notre-Dame de Paris, telle que vous l'avez connue, telle que des générations et des générations l'ont connue, parfois même sans l'avoir visitée. En dépit de nos différences, en dépit des multiples transformations architecturales que la cathédrale a connues au fil des siècles, nous en avons tous, dans notre inconscient, peu ou prou la même image.

il tient lieu d'exception ! Bref, je vous invite à aller au fond : au fond de votre mémoire rétinienne, au fond de ce que Notre-Dame de Paris représente pour toutes et tous, au fond de ce que chacun d'entre nous a ressenti lors du terrible incendie qui a sérieusement endommagé endommagé ce symbole parmi les symboles de notre culture et de notre imaginaire quotidien. D'ailleurs, ce symbole aurait été totalement détruit sans l'intervention à la fois héroïque et méthodique de nos forces de sécurité civile.

lors, essayons aujourd'hui de ne pas jouer, une fois de plus, la bataille des Anciens et des Modernes ; cessons de soupçonner la République et son Président d'arrière-pensées malignes, qui viseraient à détruire l'esprit et le sens de notre patrimoine national au nom de desseins prétendument hubristiques. Chacun autour de nous, qu'il soit chrétien ou non, a envie de voir renaître au plus vite Notre-Dame et d'agir- excusez cette expression un peu inconvenante en pareilles circonstances -sans jouer avec le feu.

Depuis 850 ans, Notre-Dame n'est pas restée en l'état. Au XIX siècle, quand Viollet-le-Duc pose cette flèche, qui s'est effondrée l'autre jour, c'est un scandale de modernité. Notre-Dame a toujours su accueillir la modernité, et c'est important, salutaire, souhaitable que d'accueillir la modernité, y compris dans l'art ou dans le travail des artisans. « Si vous regardez ce qu'il reste de Notre-Dame de Paris, l'image phare est cette statue de la Pietà du XVIII siècle, au fond du choeur, avec cette grande croix dorée au-dessus. « La grande croix, elle, a été installée en 1994. Notre-Dame a toujours su accueillir la modernité, et c'est nécessaire. « C'est une modernité qui a toujours respecté l'histoire du lieu, son passé, et surtout sa nature. »

Non, son auteur est Philippine de Saint-Pierre, directrice générale de KTO, la chaîne de télévision catholique qui a retransmis en direct, le 15 juin dernier, la première messe célébrée à Notre-Dame après l'incendie du 15 avril.

peut et doit s'opérer. Cela étant, revenons-en, ou plutôt venons-en à la version du texte de loi qui nous est proposée aujourd'hui. Les critiques au Sénat en première lecture ont été rudes et parfois violentes, jouant à l'envi de l'expression « loi d'exception »,

pour sa part, précise que les assouplissements donnés aux législations en vigueur seront strictement proportionnés aux besoins du chantier. La transparence dans le suivi de la souscription à l'égard tant du Parlement que du public et l'application du dispositif fiscal y afférent ont été renforcés. L'affectation des fonds respectera à la lettre les principes de la loi de 1905 relative à la laïcité et ceux de la loi de 1907 concernant les prérogatives respectives de l'État et des diocèses. Il y a là, je crois, pour tout esprit constructif, voire restaurateur, matière à satisfaction.

Madame la présidente, monsieur le ministre, mes chers collègues, dans quelques jours, il y aura trois mois que s'affairent, autour de la cathédrale incendiée, les personnels de la direction régionale des affaires culturelles,

Je tiens à saluer, avec la plus grande solennité, leur dévouement et leur engagement absolus au service de l'intérêt général.

Leur action exemplaire le montre bien : il est utile, et même indispensable, pour l'État et le ministère de la culture de disposer de services déconcentrés capables d'agir au plus près du terrain, dans le cadre de processus rigoureux, mais ajustables à leurs spécificités. L'ampleur remarquable et l'efficacité incontestable de cette mobilisation prouvent la qualité et l'utilité intrinsèques de la législation patrimoniale et des moyens de sa mise en oeuvre. Malgré le caractère exceptionnel du sinistre, nous n'avons pas eu connaissance d'un quelconque obstacle administratif ayant entravé les travaux. Face à l'analyse objective de ces trois mois de chantier, pourquoi modifier radicalement leur organisation ? Pourquoi bâtir une nouvelle structure sans nous expliquer pourquoi celles qui oeuvrent aujourd'hui seraient défaillantes ? Pourquoi prendre le risque d'expérimenter, dans l'urgence, de nouvelles procédures sans dresser le bilan de l'efficacité de celles appliquées maintenant ? Sans réponse précise à ces questions, nous continuerons de penser que le présent texte répond non pas aux nécessités du terrain, mais à la volonté présidentielle d'intervenir directement dans la gestion d'un chantier considéré comme un fait symbolique de la geste du quinquennat. Ce qui manque aujourd'hui à celles et ceux qui se relaient au chevet de la cathédrale, ce n'est pas une nouvelle strate administrative ; c'est, tout d'abord, le renforcement des capacités d'intervention du ministère de la culture. Ainsi, Ainsi, la quasi-totalité des moyens humains du laboratoire de recherche des monuments historiques est engagée sur le chantier de Notre-Dame. Cet effort est néanmoins insuffisant. Surtout, il prive d'une expertise indispensable toutes les autres opérations engagées ou à venir.

lors de la première lecture de ce texte, je vous avais alerté sur la nécessité d'accroître les ressources de vos services spécialisés : ils vont accompagner l'opération de restauration de la cathédrale dans la longue durée, et il serait de mauvaise politique de développer les mêmes compétences dans une nouvelle structure. L'État souhaite élever au rang d'exemple,, la réhabilitation de Notre-Dame. Il se doit donc d'être lui-même exemplaire dans son engagement budgétaire en faveur de ses services et des programmes qui vont contribuer à ce travail. Il doit nécessairement participer financièrement à cette mobilisation générale et ne pas tout attendre de l'évergétisme de généreux donateurs. Sur ce sujet, comme pour la création du centre national de la musique, dont nous avons débattu hier, nous attendons de votre ministère des engagements chiffrés lors de la discussion du projet de loi de finances pour 2020. Dans le même esprit, je vous redis l'impérieuse exigence de préparer un programme de recherche sur le monument et son environnement historique dans la longue durée, afin d'organiser les nombreuses initiatives et propositions des chercheurs français et étrangers. Il faut assurer la coordination interministérielle de ces études et leurs interactions avec le maître d'ouvrage de la restauration, sans les confondre dans la même structure, afin de garantir la destination des dons. sans attendre les résultats de l'enquête en cours, il convient d'engager une grande mission sur la protection des monuments historiques contre les risques d'incendie. Des défaillances ont été identifiées. Un diagnostic global doit être lancé. Par ailleurs, l'incendie de Notre-Dame a fait apparaître certaines lacunes de la documentation disponible sur ce monument insigne. Ainsi, la charpente avait été très peu étudiée, et il est regrettable de devoir entreprendre maintenant des analyses sur ses restes carbonisés. Cette expérience malheureuse nous oblige donc à nous interroger sur la complétude des dossiers documentaires disponibles sur nos grands édifices. « À quelque chose malheur est bon », dit l'adage populaire. Nous espérons que l'incendie de la cathédrale sera le moment d'une prise de conscience collective de l'importance des monuments historiques au sein de la cité, de leur fragilité et de l'urgente nécessité de consacrer en priorité les moyens de la Nation à leur connaissance et à leur restauration ! Bravo ! La parole

Sur le fond, la mobilisation de la société, des experts, des amoureux du patrimoine et des parlementaires a infléchi ce projet

l'environnement, ce n'est pas que des mots. On peut dire, « le réchauffement climatique, c'est dramatique, l'environnement c'est important »,

Au sein de la chambre haute, nous avons été soucieux de défendre une position commune. Dans le cadre de nos travaux en première lecture, nous avons exprimé des préoccupations susceptibles de nous réunir. Tout d'abord, nous avons refusé que ce projet de loi, qui a vocation à permettre la restauration de Notre-Dame après le sinistre du 15 avril dernier, soit un catalogue de mesures d'exception. Rien ne le justifie Monsieur le ministre, s'il existe un impératif réel qui motive vos intentions, et qui ne soit pas la seule parole présidentielle, nous vous invitons de nouveau à le porter à notre connaissance. Le monde du patrimoine, dans sa plus grande diversité, a fait part de son inquiétude devant votre empressement et devant la volonté de l'exécutif de déroger aux règles qui régissent la restauration de nos monuments historiques. La cathédrale de Paris n'a pas été édifiée pour servir le culte de l'immédiateté qui caractérise notre époque. Le Sénat a, en outre, estimé qu'il était absurde de s'employer à fixer des règles pour vouloir ensuite s'en affranchir sans motif impérieux. La restauration de cet édifice doit se faire dans le cadre commun, celui-là même que nous demandons à tous les élus et à tous les propriétaires de France de respecter lorsqu'ils entreprennent des projets de restauration. Même si Notre-Dame de Paris représente un des édifices les plus remarquables de notre patrimoine architectural, elle en demeure un élément. Si les réglementations et les normes existent, c'est qu'elles sont fondées ; sinon, proposons leur suppression

qui contenait l'essentiel des mesures d'exception. En nouvelle lecture, nous souhaitons accompagner la position de notre rapporteur, qui demeure soucieux d'oeuvrer à l'établissement d'un texte de compromis. Aussi, nous ne nous déposerons pas en séance un amendement similaire. Le Gouvernement a revu la rédaction de l'article 9 du projet de loi. Les modifications qui y ont été apportées par notre commission, sur proposition de notre collège Alain Schmitz, ont conduit à la suppression des principales mesures dérogatoires. Il s'agit là d'une nouvelle position de sagesse du Sénat et d'une main tendue à nos collègues députés, pour que nous ne donnions pas aux Français l'image d'une représentation nationale divisée sur un sujet qui devrait, au contraire, nous rassembler. demeure toutefois dans ce texte à laquelle les élus du groupe du RDSE ne peuvent toujours pas souscrire : la majoration de la déduction fiscale à 75 % consentie aux donateurs jusqu'à 1 000 euros, dont nous continuerons à demander la suppression.

Tout d'abord, cette majoration ne paraît pas se justifier, au vu de la mobilisation financière aussi spontanée que massive qui a suivi le sinistre, alors que les deniers publics font aujourd'hui très largement défaut ailleurs. Monsieur le ministre, nous avons entendu vos avertissements quant à la relative lenteur avec laquelle se concrétisent les promesses. Il n'aura cependant échappé à personne que plusieurs personnalités et de grandes entreprises ont formulé, publiquement, des promesses de dons particulièrement généreuses, dont on imagine difficilement qu'elles ne se concrétisent Monsieur le ministre, il est dans ce pays des défis qui suscitent beaucoup plus d'inquiétudes quant à notre capacité à réunir les fonds nécessaires pour les relever que celui de la restauration de la cathédrale de Paris ! En outre, même si Notre-Dame était le monument le plus visité de France et d'Europe il y a encore trois mois, il n'en demeure pas moins que nos routes et nos communes abritent des merveilles architecturales qui participent également de notre richesse nationale. nombre de ces éléments patrimoniaux sont aujourd'hui menacés et pourraient légitimement revendiquer un traitement fiscal identique. C'est vrai ! Ils auront droit au loto ... Enfin, cette majoration s'appliquant à une simple déduction d'impôt, et non à un crédit, elle exclut, de fait, la moitié de la population. Une partie des Français pourra donc faire oeuvre de générosité dans le cadre de la restauration de Notre-Dame en bénéficiant d'un accompagnement de l'État, quand l'autre ne le pourra pas. On nous oppose la parole présidentielle et celle de l'exécutif pour justifier l'impossibilité de revenir sur cette mesure, mais si le Gouvernement a jugé opportun d'annoncer, dès le lendemain du sinistre, cette majoration, ses mots n'engagent pas pour autant la représentation nationale.

Une nouvelle fois, le Sénat est soucieux de ne pas produire une loi d'exception ; un discours prônant la dérogation au règlement sous prétexte de fiabilité, voire d'efficacité, serait tout simplement inaudible. Après l'immense émotion suscitée par son incendie, la restauration de Notre-Dame de Paris ne saurait être une vitrine politique pour qui que ce soit ; elle doit être un sujet de concorde.

Il était donc tout à fait normal, compréhensible et légitime qu'il passe par la toise de l'expérience et de la réflexion des députés et des sénateurs pour atteindre sa juste et bonne mesure législative. Dans cet esprit constructif, le Sénat avait proposé en première lecture, grâce au travail du rapporteur Alain Schmitz, des corrections au texte de l'Assemblée nationale, allant dans le sens d'une plus grande cohérence dans la mise en place des dispositifs à prévoir pour la conservation et la restauration

Après cette annonce, aucun débat n'était possible et la discussion sur les autres articles devenait inutile. Par souci de convivialité, et puisque l'on nous avait annoncé que l'article 9 serait, en tout état de cause, rétabli par l'Assemblée nationale,

des mesures sur la publicité et de l'occupation du domaine public par des activités économiques, nous sommes favorables à votre texte. En revanche, nous pensons qu'il ne faut pas supprimer la consultation de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture,

Si nous saluons le fait que vous ne proposiez plus de dérogation au code du patrimoine, vous maintenez cependant le principe d'une dérogation par ordonnances aux codes de l'environnement, de la voirie et de l'urbanisme,

de la date d'entrée en application de la déductibilité fiscale. De nombreux dons ont été effectués le 15 avril, dans l'intention de contribuer à la restauration de Notre-Dame. Ce n'est pas parce que le Président de la République a dit : « dès demain ... » qu'il faut, par la loi, instaurer par la loi, instaurer une inégalité de traitement entre ceux qui ont versé le 15 et ceux qui ont donné le 16. Comme vous le savez, monsieur le ministre, mes chers collègues, nous restons, comme nombre de Français et beaucoup de donateurs, désireux de voir la cathédrale et sa flèche reconstruites dans le dernier état visuel connu.

De très nombreux monuments historiques prestigieux de Paris en sont couverts, sans que cela gêne le moins du monde ; c'est le cas du dôme du Panthéon, du dôme des Invalides, de la toiture de la flèche de la Sainte Chapelle, construite en bois et recouverte de plomb, et de bien d'autres monuments historiques de Paris. Et le Sénat ? Je me permets, enfin, de rappeler que la toiture du château de Versailles a été restaurée au plomb. Nous nous réjouissons que vous ayez tranché l'ambiguïté que contenait le texte initial à l'article 8 et que vous ayez clairement opté pour un établissement public à caractère administratif, placé sous l'autorité du ministre de la culture pour la maîtrise d'ouvrage des opérations. Nous tenons cependant à ce qu'il soit précisé que la maîtrise d'oeuvre sera assurée sous l'autorité de l'architecte en chef des monuments historiques.

je puis témoigner de l'intérêt tout particulier exprimé par ses membres à l'exposé de M. l'architecte en chef des monuments historiques, Philippe Villeneuve, sur l'état des lieux détaillé au lendemain de l'incendie et sur toutes les mesures prises au titre de l'urgence.

La CNPA a pris acte de la précarité de la situation et de la fragilité des structures de l'édifice, impliquant la nécessité d'achever les travaux de sécurisation et de consolidation qui ont été

J'espère que cette séance, au cours de laquelle nous allons pouvoir constater de nombreux points de convergence entre l'Assemblée nationale et le Sénat, verra également quelques-unes de nos propositions acceptées et incluses dans le texte qui deviendra

En nouvelle lecture, l'Assemblée nationale a rétabli son texte de première lecture, avec un bémol a précisé que les fonds de la souscription seraient exclusivement destinés au financement des travaux de conservation et de restauration de la cathédrale et de son mobilier, ainsi qu'à la formation de professionnels.

incohérent. Ainsi, l'article 8 prévoit que l'établissement public ayant pour mission d'assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations pour la conservation et la restauration de la cathédrale pourra réaliser l'aménagement de l'environnement immédiat de la cathédrale et mettre en oeuvre, avec les ministères concernés, des actions culturelles et éducatives de valorisation des travaux. Cette préoccupation rejoint la nôtre, mais nous nous interrogeons sur le mode de financement qui sera retenu, puisque, désormais, le produit de la souscription sera

d'autres fins que la restauration de la cathédrale et de son mobilier, dont l'État est propriétaire, et la formation des compétences requises pour le chantier. Vous souhaitez notamment pouvoir étendre le périmètre du financement à l'aménagement des abords de la cathédrale, compte tenu de l'extension du périmètre d'intervention de l'établissement public. C'est malheureusement juridiquement impossible, puisque les organismes collecteurs chargés de recueillir les dons dans le cadre de la souscription, en particulier les fondations reconnues d'utilité publique, sont dotés d'un statut de droit privé et ont l'obligation de respecter l'intention des donateurs. Or il n'a jamais été question, au moment où ceux-ci ont versé leur don, que le champ de la souscription ne porte pas exclusivement sur la restauration de la cathédrale consécutivement au sinistre.

Il s'agit de revenir à la rédaction initiale, plus simple et plus claire, fondée sur l'intérêt historique, artistique et architectural du monument.

plus d'un siècle d'organiser des débats rationnels et structurés sur la nécessité de restaurer ou de ne pas restaurer et de le faire de façon plus ou moins fidèle.

revient pas au législateur de définir un choix esthétique. Mais dans ce cas, nous aurions dû commencer par discuter de l'article 9 et le supprimer

des dons, notamment pour les objets mobiliers qui sont dans Notre-Dame de Paris et qui nécessitent une restauration.

ignoraient, au moment où ils ont versé leurs dons, que cette somme pourrait être utilisée pour une autre finalité que la restauration de la cathédrale. Ouvrir cette possibilité créerait donc un risque juridique.

l'État propose, au travers de cette rédaction, que l'établissement public puisse bénéficier d'une délégation de maîtrise d'ouvrage afin d'effectuer les travaux dans le cadre d'un financement à déterminer.

d'aménagement de l'environnement immédiat de Notre-Dame de Paris. Franchement, je ne vois pas où est le problème. Le Gouvernement

le bien, c'était l'Hôtel-Dieu ; et le vrai- chacun trouvera sa vérité -, c'était l'école cathédrale.

L'enjeu est de savoir quels moyens l'État doit consentir pour accompagner le chantier tout en respectant la priorité de donation des dons.

des finances lors de la nouvelle lecture, avant d'être réintroduite en séance publique. À nos yeux, cette majoration ne se justifie toujours pas, compte tenu de la mobilisation financière aussi spontanée que massive entourant le sinistre, alors que les deniers publics font largement défaut ailleurs. Par ailleurs, cette majoration s'applique à une déduction d'impôt et non à un crédit, ce qui exclut de fait la moitié de la population. Si le Gouvernement a jugé opportun d'annoncer

; c'est une bonne chose, car il aurait été critiqué, et à juste titre, s'il n'avait pas été présent dès le 15 avril au soir et s'il n'avait pas souhaité agir au plus haut niveau de l'État

Je comprends l'amendement de Mme Jouve, mais le Président de la République s'était engagé à mettre en place une défiscalisation à hauteur de 75 %. Quand un engagement est pris et que les dons se font sur cette base, il est très compliqué, comme l'a souligné le rapporteur, de revenir en arrière, même si, fondamentalement, pour ma part

Vous le savez, nos concitoyens les plus démunis ne payent pas d'impôt sur le revenu. Ce dispositif d'encouragement fiscal s'adressera à tous, sauf à ceux qui ont peu de revenus,

proposée se justifie pour renvoyer à la clarification des conditions dans lesquelles le produit de la souscription peut être reversé, soit à l'établissement public, soit à l'État, que nous avons introduite à l'article 3 du projet de loi. C'est pourquoi

a pour objet de clarifier les missions de l'établissement public d'État désigné pour la reconstruction de Notre-Dame de Paris en matière de maîtrise d'ouvrage déléguée. Je rappelle que le maître d'ouvrage est l'entité porteuse du besoin, définissant l'objectif du projet, son calendrier, etc. Le résultat attendu du projet est la réalisation d'un produit, c'est-à-dire l'ouvrage. Le maître d'oeuvre, lui, est l'entité retenue par le maître d'ouvrage pour réaliser l'ouvrage dans les conditions de délai, de qualité et de coût fixées par ce La maîtrise d'oeuvre est donc responsable des choix techniques inhérents à la réalisation de l'ouvrage, conformément aux exigences de la maîtrise d'ouvrage. Le texte exigences de la maîtrise d'ouvrage. Le texte charge l'établissement public « d'assurer la conduite, la coordination et la réalisation des études et des opérations » de conservation et de restauration. Cette rédaction procède ainsi à un mélange des genres entre ce qui relève de la maîtrise d'ouvrage et de la maîtrise d'oeuvre. Nous voulons limiter clairement le rôle de l'établissement public à la maîtrise d'ouvrage, c'est-à-dire le rôle pour lequel il est créé.

Nous avons rétabli en commission la disposition que nous avions adoptée en première lecture pour garantir- c'est un point essentiel -que la maîtrise d'oeuvre resterait exercée sous l'autorité de l'architecte en chef des monuments historiques.

vise à supprimer la référence aux compétences de l'architecte en chef des monuments historiques, à la composition du conseil scientifique et aux précisions relatives à la dissolution de l'établissement public, et à réintroduire la dérogation relative à la limite d'âge. d'âge. La compétence de l'architecte en chef des monuments historiques est prévue par la partie réglementaire du code du patrimoine. La composition du conseil scientifique relèvera du décret.

parole est à M. le rapporteur. Cet amendement vise à préciser les zones dans lesquelles l'établissement public pourrait être chargé de conduire des travaux d'aménagement pour mettre en valeur et améliorer les accès de la cathédrale de Paris.

Nous proposons, par conséquent, que soient bien explicitées les zones concernées, à savoir le parvis, les deux squares entourant la cathédrale et la promenade du flanc sud de l'île de la Cité, c'est-à-dire celui qui longe les berges de la Seine. Pour ne rien vous cacher, il s'agit des zones qui étaient mentionnées dans l'exposé des motifs de l'amendement que le Gouvernement avait déposé à l'article 8 à l'Assemblée nationale en nouvelle lecture. La commission a décidé tardivement de déposer cet amendement, pour opérer une coordination avec l'amendement déposé par Mme Vérien à l'article 9, qui tend à préciser de la même manière les zones susceptibles de faire l'objet de travaux d'aménagement.

Le risque serait grand de voir le Gouvernement lui demander, une fois les travaux de restauration achevés, de se substituer à l'État pour assurer son entretien courant. Néanmoins, il est difficile de prévoir une date fixe de la durée de vie de cet établissement public, compte tenu compte tenu des incertitudes qui pèsent encore sur l'état de la cathédrale et sur le temps nécessaire pour la restaurer, au regard de tous les aléas qui peuvent affecter un chantier. Nous souhaitons, par notre amendement, prévoir que la durée d'existence de l'établissement public sera celle des travaux directement induits par l'incendie

pour toute la durée du chantier. Il s'agit donc d'un usage

a un instant notre position sur la question de la maîtrise d'oeuvre, et il s'agit d'un point essentiel pour nous. Vous reconnaissez vouloir faire figurer dans la loi des dispositions qui ne sont pas nécessaires, comme la dérogation à la limite d'âge, rendue de toute façon possible en vertu d'une loi en vigueur. C'est pour cette raison que nous voulions sécuriser les choses sur la maîtrise d'oeuvre et la maîtrise d'ouvrage. la dérogation à la limite d'âge, la commission a estimé lundi dernier qu'il s'agissait d'une question de principe ; nous ne souhaitons pas nous associer à l'idée d'une loi d'exception. Enfin, nous estimons important que l'établissement public soit dissous au terme de l'achèvement des différents travaux dont il a la charge. C'est pourquoi nous avons précisé les grands principes qui devraient être mis en oeuvre par le décret relatif à la dissolution de l'établissement. La commission émet donc un avis défavorable sur l'amendement présenté par le Gouvernement.

C'est pourquoi le texte de commission prévoit un grand principe sur les circonstances de la dissolution, sans remettre en cause la nécessité d'un décret, pour en préciser les modalités exactes d'application. C'est la raison pour laquelle, monsieur Assouline, je vous propose

permet d'encadrer suffisamment la compétence de l'établissement public. Si le parvis et les squares entourant la cathédrale et la promenade du flanc sud de l'île de la Cité font effectivement partie de cet environnement immédiat, comme je l'ai d'ailleurs précisé dans mon discours, les espaces contigus à ces lieux pourraient devoir être inclus dans les travaux. Il faut se laisser une petite marge de manoeuvre.

compte tenu du caractère de trésor national que revêt Notre-Dame de Paris, de son insertion dans un site inscrit au patrimoine mondial de l'Unesco et du caractère délicat des travaux qui devront être mis en oeuvre pour sa conservation et sa reconstruction. Il est surprenant de constater que le Gouvernement n'a pris qu'à moitié la mesure de nos remarques, des remarques des experts et des conservateurs de musée, comme vient de le dire M. Ouzoulias, et qu'il recoure aux ordonnances pour déroger à de très nombreux textes législatifs. Désormais, le projet de loi prévoit directement certaines de ces dérogations, mais mais procède par ordonnance pour en fixer d'autres. Concernant les dérogations désormais prévues aux termes de ce texte, il est aberrant de prévoir que, le cas échéant, l'établissement public se substituera à un opérateur de fouilles archéologiques bénéficiant d'un agrément de l'État, surtout si celui-ci sous-traite à l'Inrap,

elle n'est pas acceptable, et je me réjouis de sa suppression par notre commission. Cette dérogation donnait encore un coup de canif aux avis des ABF et créait un précédent fâcheux en termes de protection des monuments

Il a partiellement entendu le message que nous avions adressé lors de la première lecture : nous avions alors jugé inacceptable la mise en place de dérogations susceptibles de couvrir un périmètre très large- j'allais dire trop large -et de mettre en danger notre législation en matière de patrimoine. Vous nous l'avez redit, monsieur le ministre, vous avez circonscrit le champ des dérogations au code du patrimoine, au code général de la propriété des personnes publiques et aux règles de publicité prévues par le code de l'environnement, en indiquant précisément- ce que nous avions souhaité -les dérogations concernées. Vous avez par ailleurs exclu les règles de la commande publique du champ des dérogations. nous avons supprimé l'habilitation à déroger par ordonnances aux règles en matière de voirie, d'environnement et d'urbanisme, ainsi qu'aux règles applicables aux travaux et aux aménagements et constructions utiles pour ces travaux.

dispense de consultation de la commission régionale du patrimoine et de l'architecture, la CRPA, car elle aurait pu créer un précédent dangereux en matière de protection du patrimoine. Dans ces conditions, et eu égard aux efforts tout à fait considérables que le Gouvernement a consentis à la Haute Assemblée, il ne me paraît pas souhaitable de rejeter en bloc l'article 9, dont une partie des dispositions pourraient simplifier la mise en oeuvre du chantier et sa valorisation. du chantier et sa valorisation. Le principe d'une interdiction de la publicité a été clairement posé par le Gouvernement, notamment sur les bâches de chantier. Les seules publicités autorisées sur ces bâches, sur les palissades situées aux abords de la cathédrale et sur les installations provisoires ou définitives situées dans l'emprise du chantier sont celles qui ne présenteront pas de caractère commercial et qui viseront exclusivement à informer le public sur les travaux, et à mettre en valeur, ce qui me semble essentiel, la formation initiale et continue des professionnels

que vous avez réalisé, monsieur le ministre, pour en circonscrire le champ et indiquer précisément dans la loi celles qui concerneraient le code du patrimoine, le code général de la propriété des personnes publiques et les règles de publicité prévues par le code de l'environnement. Toutefois, comme je l'ai déjà indiqué, la dispense de consultation de la CRPA nous semble particulièrement problématique en ce qu'elle fait que le préfet de région est dans cette affaire à la fois juge et partie. Par ailleurs, compte tenu du manque de motivation de votre demande d'habilitation et du manque de précision sur la nature et le champ des dérogations susceptibles d'être concernées, nous ne pouvons pas y souscrire.

Le délai de quinze jours proposé par Mme Vérien me paraît intenable. Cela créerait par ailleurs un précédent extrêmement dangereux à l'avenir : en effet, pourquoi autoriser à raccourcir les délais pour le chantier de Notre-Dame de Paris et pas pour n'importe quel autre projet de restauration ? Là encore, cela me semble être une dérogation dangereuse. C'est pourquoi la commission a émis un avis défavorable

Néanmoins, nous ne sommes toujours pas satisfaits de ce texte, dont nous ne comprenons toujours pas l'utilité juridique et opérationnelle. On en comprend bien l'utilité politique, mais, encore une fois, mes chers collègues, la transposition législative de la parole présidentielle n'est pas un argument dirimant nous. Nous voterons contre ce texte, parce que l'on peut s'en passer et continuer à travailler sur le chantier de la restauration comme tous les personnels de la culture le font, de façon admirable, en ce moment. Ces derniers n'ont pas besoin de ce texte de loi, mais d'un soutien fort de leur ministère, qui leur manque sensiblement en ce moment. Je n'ai aucune illusion sur l'issue du vote, mais je crois qu'il est très important, madame la présidente de la commission, que, dans la tradition de cette assemblée, nous suivions de façon très ferme et très précisément la manière dont cette loi loi sera mise en oeuvre sur le terrain. Il est important que notre commission puisse avoir accès à la totalité du

par le Sénat et l'Assemblée sur le projet de loi pour la conservation et la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris et instituant une souscription nationale à cet effet. Ce sujet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

Vous êtes aujourd'hui sur le point de l'adopter définitivement. Je tiens d'abord à saluer la ténacité des sénateurs Thani Mohamed Soilihi et André Reichardt, qui illustre combien la simplification, notamment lorsqu'elle porte sur des sujets très techniques, est un travail de longue haleine et doit être constamment poursuivie. de loi a su évoluer grâce au débat parlementaire : vous l'avez modifié, puis nous avons tiré ensemble les conséquences des lois adoptées depuis son dépôt, puisque certains articles étaient devenus sans objet ou étaient satisfaits la croissance et la transformation des entreprises, dont cette proposition de loi est un prolongement naturel, car elle va dans le sens de la simplification pour les entreprises. Comme vous le savez, la simplification de la vie des entreprises est au coeur de l'action que nous menons au ministère de l'économie.

Cela doit également être un axe structurant de notre action sur le plan réglementaire, tant pour les PME-TPE que pour l'industrie. L'objectif principal de tous ces dispositifs est de permettre à nos entreprises de pouvoir concentrer leur énergie sur le plus important : leur activité, leur croissance et la création de nouveaux emplois. La proposition de loi que nous examinons aujourd'hui s'inscrit dans cet esprit. Elle prévoit des ajustements techniques qui permettront de simplifier et de clarifier le code de commerce. Les députés, de leur côté, ont adopté des modifications utiles pour améliorer certains articles du texte en prenant en considération les positions exprimées par les sénateurs,

Il est regrettable qu'il ait fallu attendre si longtemps pour voir ce texte aboutir, car dès l'origine tout le monde s'accordait à reconnaître la pertinence et l'urgence des mesures proposées par notre collègue, dans le prolongement des travaux qu'il avait conduits en tant que rapporteur de la commission des lois du Sénat sur la loi du 2 janvier 2014. C'est tellement vrai qu'un grand nombre de ces dispositions ont été reprises, souvent à l'identique, dans plusieurs véhicules législatifs intervenus depuis : citons,

de loi a donc connu des évolutions très sensibles depuis son dépôt il y a près de cinq ans, car il a fallu en retirer les dispositions reprises dans différents textes, en actualiser d'autres, mais aussi introduire de nouvelles mesures visant à répondre aux besoins les plus récents exprimés par les professionnels, ou même à corriger à corriger les malfaçons introduites par d'autres textes. Cette proposition de loi répond à un objectif consensuel, à savoir simplifier l'environnement juridique de nos entreprises pour renforcer leur compétitivité, mais sans mettre à mal le principe de sécurité juridique. C'est ce qui explique que les deux assemblées aient fait preuve jusqu'à présent d'une très large convergence de vues. En première lecture, nos collègues députés n'ont apporté au texte que des modifications légères et, pour la plupart, tout à fait bienvenues. Il subsiste quelques points de désaccord, sur lesquels je vais revenir dans un instant. mes chers collègues, la description complète des dispositions contenues dans ce texte qui figure dans le rapport écrit. Je vous rappellerai seulement que ces mesures se répartissent en trois catégories : premièrement, la simplification de règles de fond ou de forme applicables aux actes des sociétés civiles et commerciales et des autres commerçants ; deuxièmement, l'allégement des sanctions civiles encourues lorsqu'un acte a été pris en méconnaissance des règles qui lui sont applicables ; troisièmement, la la clarification de certaines dispositions légales. Je vous propose d'examiner chacune de ces trois catégories, en commençant par la simplification des règles de fond ou de forme. Tous les Tous les actes des entreprises, en particulier ceux des entreprises qui sont exploitées sous la forme sociétaire, sont naturellement soumis à des règles de fond et de forme visant à garantir les droits des associés, des salariés, des créanciers, des parties aux autres contrats passés par la société ou l'entrepreneur, ou encore des tiers. C'est bien sûr légitime et nécessaire. Encore faut-il conserver à l'esprit que ces règles, singulièrement lorsqu'elles imposent l'accomplissement de longues formalités pour des actes courants, ont un coût pour nos entreprises, et qu'elles sont susceptibles de faire fuir les investisseurs si elles sont plus contraignantes que celles des pays voisins. Ces règles doivent donc être strictement proportionnées à l'objectif poursuivi. Prenons un exemple. depuis 1935 -, l'acte de cession d'un fonds de commerce doit obligatoirement comporter un certain nombre de mentions de mentions : le nom du précédent vendeur du fonds, ainsi que la date et le prix de la précédente cession, l'état des privilèges et nantissements grevant le fonds, le chiffre d'affaires et le résultat d'exploitation des trois exercices précédents, mais aussi, le cas échéant, les caractéristiques du bail commercial. Ouf ! À défaut, le cessionnaire peut demander au juge l'annulation de la cession, ce qui nourrit un abondant contentieux. Or, en pratique, l'acquéreur d'un fonds de commerce est un professionnel- on peut l'espérer -, qui s'entoure des services d'autres professionnels- on peut l'espérer -pour réaliser la cession, afin d'obtenir l'ensemble des informations dont il a besoin pour former son jugement. En outre, les mentions légales obligatoires ne comportent pas l'ensemble des informations nécessaires pour apprécier la valeur du fonds.

générale des actionnaires d'une société anonyme un projet d'augmentation du capital réservée aux salariés. Le renforcement de l'actionnariat salarié est naturellement un objectif louable et largement partagé. Toutefois, cette obligation triennale s'est révélée parfaitement inefficace pour atteindre cet objectif. Les sociétés qui souhaitent développer l'actionnariat salarié n'attendent évidemment pas ces rendez-vous obligatoires qui, ailleurs, se révèlent purement formels. Je suis donc particulièrement satisfait que l'Assemblée nationale ait adopté conforme l'article 27 de la proposition de loi, qui vise à supprimer cette formalité. Examinons maintenant la question de l'allégement des sanctions civiles. Les actes pris en méconnaissance des règles légales s'exposent à de telles sanctions. La sanction la plus lourde est la nullité de l'acte, qui peut être obligatoire ou facultative, c'est-à-dire laissée à l'appréciation du juge, absolue ou relative, autrement dit susceptible d'être invoquée par la seule partie protégée. Dans certains cas, cette sanction peut être avantageusement remplacée, à mon avis, par une injonction de faire : plutôt que d'annuler l'acte entaché d'irrégularité, le juge enjoindra à la société ou à l'entrepreneur de remplir ses obligations, ce qui couvrira l'irrégularité. il est indispensable que la sanction civile soit proportionnée à l'objectif poursuivi, car le risque d'annulation est un facteur d'insécurité juridique pour toutes les parties. Je me félicite donc que les députés aient adopté conforme l'article 26, qui remplace la nullité obligatoire des délibérations adoptées par l'assemblée générale d'une société anonyme sans avoir été inscrites à l'ordre du jour par une nullité facultative, qui laisse au juge un pouvoir d'appréciation.

qui visait à remplacer par une injonction de faire la sanction de nullité obligatoire frappant les décisions d'augmentation de capital prises en méconnaissance de l'obligation légale de soumettre simultanément à l'assemblée générale un projet d'augmentation de capital réservée aux salariés. Une injonction de faire serait pourtant une sanction beaucoup plus adaptée. Je note d'ailleurs que la jurisprudence la plus récente de la Cour de cassation nous donne raison, puisqu'elle admet désormais qu'une augmentation de capital irrégulière puisse être régularisée par le vote ultérieur, même négatif, sur un projet de résolution réservant une augmentation de capital aux salariés.

Ces mesures de clarification sont, pour certaines d'entre elles, attendues depuis des années, voire des décennies- n'est-ce pas, cher Thani Mohamed Soilihi ? -, comme celle qui concerne les droits

D'autres dispositions tendent à clarifier des mesures qui viennent tout juste d'être introduites dans notre droit, à l'occasion de la loi Pacte, par exemple les conditions dans lesquelles une minorité d'associés peut obtenir la nomination d'un commissaire aux comptes, à l'article 54 . Je veux dire un mot des dispositions relatives aux commissaires aux comptes, qui constituent le chapitre IV de cette proposition Nous avons été sollicités, en vue de cette deuxième lecture, par des commissaires aux comptes et par d'autres professionnels- n'est-ce pas, monsieur le président de la commission des lois ? -qui s'inquiètent des conséquences de la loi Pacte. loi a procédé à une importante réforme des missions des commissaires aux comptes. Dans l'ensemble, cette réforme a recueilli l'assentiment du Sénat, car un équilibre a été trouvé entre des impératifs et des intérêts partiellement

nous serons attentifs à la mise en oeuvre de cette réforme, et nous serions heureux que le Gouvernement nous fasse part de ses intentions en ce qui concerne la révision du code de déontologie des commissaires aux comptes, qui nous paraît une problématique paraît une problématique à prendre en compte rapidement. Je dois dire que nous avons été surpris de voir introduire par voie d'amendement, à l'Assemblée nationale, une disposition visant à lever le secret professionnel des commissaires aux comptes à l'égard de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques et du juge de l'élection. Il s'agit Il s'agit à l'évidence d'un cavalier législatif. Toutefois, la commission a estimé cette mesure bienvenue sur le fond et l'a donc maintenue, car elle contribuera à la transparence de la vie politique française. française. Malgré quelques désaccords avec nos collègues députés, la commission a estimé que le texte soumis à l'examen du Sénat constituait un compromis satisfaisant. Afin de ne pas retarder une nouvelle fois, cher Thani Mohamed Soilihi,

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, nos entrepreneurs doivent faire face à bon nombre d'obstacles. L'environnent commercial de nos entreprises est de plus en plus instable, en raison notamment de la multiplication de sanctions extraterritoriales imposées par les États-Unis. Un entrepreneur français ayant une activité internationale doit sans cesse surveiller les embargos et les sanctions commerciales qui s'appliquent à plus d'une trentaine de pays, à des personnes morales et physiques, à des marchandises ou à des moyens de transport. Au quotidien, nos entreprises doivent ainsi s'assurer que leurs opérations ne sont pas visées par des sanctions qui tombent sans préavis.

C'est pourquoi les mesures inscrites dans la proposition de loi que nous examinons cet après-midi nous paraissent nécessaires et judicieuses ; elles vont dans le bon sens. Les concepteurs du code de commerce de 1807 avaient un objectif que nous devons garder en tête : la création d'un cadre juridique favorable au développement de l'activité économique. La finalité du droit est le bien commun. Lorsque la réglementation devient un fardeau, c'est que quelque chose ne va plus et qu'il faut revoir les règles.

Le texte a été mis à jour au fil des évolutions du droit intervenues depuis son dépôt. Le travail du rapporteur a mis en lumière le caractère consensuel des dispositions proposées encore en discussion. en discussion. Nous souhaitons tous ici que nos entreprises puissent se consacrer à la création de richesse sans être accaparées par la résolution de questions posées par des règles obscures et inutilement complexes. Le temps passé sur ces problématiques techniques, c'est du temps perdu, et donc, évidemment, de l'argent perdu, voire de la compétitivité en moins. Les mesures proposées vont dans le bon sens. La consultation écrite des actionnaires lors de la prise de décisions d'importance secondaire nous paraît pertinente. De même, la clarification des droits de vote en cas de démembrement d'une part de société civile est indispensable. Nous pensons que cette précision permettra d'éviter de nombreuses procédures judiciaires.

Ce processus de simplification n'est pas achevé. Il faudra continuer à oeuvrer pour sécuriser et clarifier l'environnement juridique de nos entreprises. La masse des réglementations et la complexité de certaines normes doivent nous conduire Et cette réflexion ne concerne pas que le droit des sociétés. Nous devons veiller à n'adopter que des lois nécessaires, claires et intelligibles. Pour l'heure, le groupe Les Indépendants se réjouit des mesures figurant dans la proposition de loi et votera en faveur de l'adoption Nous espérons également que la simplification sera poursuivie par le biais d'autres initiatives contribuant à favoriser le développement de nos entreprises. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi.

le présent texte avait été déposé sur le bureau du Sénat en août 2014- ça ne nous rajeunit pas ! Il avait été examiné et adopté en commission des lois le 1 juin 2016, pour n'être inscrit à l'ordre du jour de notre assemblée, dans un espace réservé au groupe La République En Marche, qu'en mars 2018. Ce n'est encore qu'un an plus tard qu'il a été discuté et adopté par nos collègues députés à l'unanimité Au cours de la discussion générale, certains ont pu s'étonner que cette proposition de loi n'ait pas été intégrée à la loi relative à la croissance et la transformation des entreprises, dite loi Pacte. La raison en est simple : je voulais une loi à mon nom Je plaisante, bien évidemment ! La loi Pacte comportait déjà 221 articles ... De plus, toutes les dispositions contenues dans ma proposition de loi n'auraient pas trouvé leur place dans ce texte, ce qui, vous en conviendrez, aurait été fort dommage. En effet, si nombre d'entre elles ont été reprises dans d'autres véhicules législatifs, tels que la loi Macron du 6 août 2015, la loi Sapin II du 9 décembre 2016 ou d'autres textes que vous avez également cités, monsieur le rapporteur,

le rapporteur. Merci, cher André, d'avoir réalisé ce fastidieux et très technique travail de dépoussiérage et d'actualisation de ce texte.

Mais je sais que les dispositions qu'elle contient permettront de répondre aux demandes exprimées par les acteurs du tissu économique.

et à tous ceux- ils sont nombreux -qui se trouvent dans une situation analogue. Pour toutes ces raisons, je suis soulagé qu'un peu de temps, après cinq années d'errance dans les méandres de la navette parlementaire, ait enfin été trouvé pour l'examen de cette proposition de loi. de loi. Nous avions, en première lecture, adopté ce texte à l'issue d'un débat qui avait duré moins de trois heures. Contrairement à une idée reçue, et comme l'avait fait remarquer à l'époque M. le ministre Bruno Le Maire, avancer à un train de sénateur signifie aller plus vite que la lumière.

J'en citerai néanmoins quelques-unes : mesures relatives au fonds de commerce- suppression des mentions légales obligatoires dans les actes de vente, facilitation et simplification du régime de la location-gérance location-gérance ; précisions apportées sur le démembrement des parts sociales ; simplification des conditions de remplacement du gérant d'une société civile en cas de vacance, d'une part, et du régime de fusion des sociétés civiles, ; création dans le code civil d'une procédure de régularisation de la prorogation d'une société au-delà de son terme normal en cas d'omission de bonne foi ; suppression de l'obligation trisannuelle de une résolution tendant à la réalisation d'une augmentation de capital réservée aux salariés, qui était inutile ; simplification de l'octroi par une société mère de cautions, avals et garanties aux sociétés qu'elle contrôle ; non-comptabilisation comme votes négatifs des abstentions et des votes blancs ou nuls des actionnaires dans les assemblées générales ; facilitation du recours à la dématérialisation des assemblées générales, tout cela parmi bien d'autres dispositions de dépoussiérage, d'actualisation et de simplification. Une chose est certaine ces mesures sont toutes attendues de pied ferme par nos entreprises ! Je serai donc bref, et ajouterai seulement, pour conclure, que je ne doute pas que nous examinerons aujourd'hui ce texte avec la même célérité. J'espère également, au nom des entreprises de notre pays, que cette proposition de loi fera, comme en première lecture et comme à l'Assemblée nationale, l'objet d'une belle unanimité. La parole

Au final, la chambre haute, en commission, ayant adopté sans modification, en seconde lecture, le texte de l'Assemblée nationale, il ne reste plus qu'à attendre la publication de celui-ci, donc à attendre encore un peu

bien qu'il soit très utile, je me contenterai de rappeler la position d'abstention de mon groupe, telle qu'elle fut d'ailleurs exprimée en première lecture.

de consentir des stock-options- je sais bien qu'il ne faut pas désespérer la City -ou aux salariés attributaires d'actions gratuites de les revendre, qui consiste, à l'article 47, à raccourcir le délai durant lequel un commissaire aux comptes ayant réalisé une mission au sein d'une société ne peut être désigné pour établir un rapport sur la création d'actions de préférence. À l'heure où l'on chasse les conflits d'intérêts, il vaut peut-être mieux, s'agissant de ce type d'opérations, Il ne nous semble pas non plus de bonne politique de supprimer l'obligation triennale de soumettre à l'assemblée générale une augmentation de capital réservée aux salariés.

Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, le groupe socialiste et républicain salue l'initiative de Thani Mohamed Soilihi, qui remonte désormais à près de cinq ans- cela a été rappelé -, ainsi que sa ténacité sa ténacité à vouloir faire adopter des dispositions qui seront utiles, à la fois parce qu'elles vont dans le sens de la simplification de plusieurs procédures et parce qu'elles favoriseront le développement de notre vie économique.

Il faut néanmoins le faire avec mesure et avec tact, car certaines procédures ont été mises en oeuvre dans le but de promouvoir une meilleure transparence de la vie économique ou de renforcer les droits des actionnaires. peuvent donc aussi constituer, parfois, des garanties utiles ; il faut y réfléchir à deux fois avant de les supprimer purement et simplement. De nombreuses dispositions ont déjà été adoptées conformes au fil de l'examen des nombreux textes portant sur des sujets économiques dont le Parlement a été saisi ces dernières années. S'agissant tout d'abord des fonds de commerce, la mesure qui tend, par l'abrogation de l'article L. 141-1 du code de commerce, à supprimer les informations qui doivent être mentionnées par le cédant dans tout acte de cession amiable d'un fonds est très utile. est nécessaire d'encourager le recours au régime de la location-gérance des fonds de commerce en supprimant la condition selon laquelle le loueur doit avoir exploité le fonds pendant deux ans. S'agissant des S'agissant des sociétés civiles, nous souhaitons saluer les dispositions qui permettent la dématérialisation des formalités de cession de parts de société civile auprès du registre du commerce et des sociétés, à l'instar de ce qui a été fait pour les SARL,

en son article 14, le remplacement du gérant d'une SARL placé en tutelle ou en curatelle. L'Assemblée nationale a restreint cet article en y excluant la curatelle, au motif qu'il serait disproportionné que la loi puisse automatiquement mettre fin

Ces modifications souhaitées par les députés nous semblent raisonnables, la curatelle étant un régime d'assistance et non de représentation. Nous saluons également la disposition visant à faciliter l'octroi par une société mère de garanties aux filiales qu'elle contrôle. L'article 21 du texte, quant à lui, met fin à une règle selon laquelle le vote d'abstention des actionnaires équivaut à un vote négatif. Il nous semble opportun que cette situation soit enfin clarifiée. Nous tenons également à saluer l'initiative, concrétisée entre-temps par voie d'ordonnance, qui offre la possibilité aux sociétés cotées de regrouper dans un document de référence unique l'ensemble des informations qu'elles sont légalement tenues de publier, comme le rapport de gestion, le rapport du président, les comptes annuels ou les données sociales et environnementales. Si l'on peut faire en sorte qu'il n'y ait plus qu'un seul document synthétique, personne ne s'en plaindra. De même, la proposition tendant à autoriser la dématérialisation des assemblées générales ordinaires des actionnaires dans les sociétés non cotées va dans le bon sens. nationale a d'ailleurs souhaité restreindre la possibilité pour des actionnaires représentant au moins 5 % du capital social de s'opposer à cette dématérialisation : ceux-ci ne pourraient exercer ce droit

Nous sommes en outre favorables à l'assouplissement des périodes d'interdiction d'attribution aux salariés de stock-options ou d'actions gratuites, afin de favoriser l'actionnariat des salariés toutes les propositions qui permettent de mieux associer les salariés au devenir de leur entreprise doivent en effet être défendues. Nous avons été particulièrement sensibles au fait que le texte initial étende la norme professionnelle simplifiée de contrôle légal des comptes aux associations et autres entités du secteur non marchand, lorsque leur total de bilan, leurs ressources ou le nombre de leurs salariés sont inférieurs à des seuils fixés par décret. Cette mesure, comme d'autres, ne fera cependant pas l'objet de nos discussions, cet article étant désormais satisfait par la loi Pacte. Mes chers collègues, je n'ai bien sûr pas fait le rappel exhaustif des dispositions figurant dans cette proposition de loi ni des apports dus à notre rapporteur, André Reichardt, au cours de la navette. J'ai en tout cas le sentiment que cette proposition de loi témoigne d'un travail détaillé et précis. Je tiens donc à féliciter notre collègue Thani Mohamed Soilihi, ses travaux aboutissant aujourd'hui à ce texte pragmatique et précieux pour l'ensemble de nos acteurs économiques. Nous voterons évidemment Pour les raisons évoquées dans mon propos introductif, il sera sans doute utile d'en faire une complète évaluation dans un délai de deux ou trois ans. Mais je ne doute pas que la commission des lois saura s'en saisir. La parole est à M.

Si la demande de stabilité juridique de la part de nos concitoyens et en particulier des agents économiques est forte, elle ne saurait réduire l'aspiration des mêmes acteurs à l'adaptation constante de notre droit. Cette adaptation régulière du droit des sociétés est un impératif pour doter nos entreprises des moyens juridiques de développer leurs activités et, en même temps, de garantir un environnement économique de confiance, qui doit être établi aussi bien à l'intérieur de l'entreprise, entre actionnaires, dirigeants, salariés, qu'à l'extérieur, à l'égard des tiers, qu'il s'agisse des clients, fournisseurs, administrations ou autres partenaires. Nous n'en sommes pas au premier texte sur le sujet. Le droit des sociétés a régulièrement évolué pour s'adapter aux mutations de l'économie, avec, parfois, certaines innovations, comme le statut simplifiée, la SAS, qui connaît un succès grandissant depuis quelques années, ou celui d'autoentrepreneur, qui, pour sa part, n'est pas concerné par le droit des sociétés, puisqu'il représente surtout une dérogation à celui-ci. On peut également noter le recours de plus en plus fréquent par les TPE, PME ou ETI aux sociétés civiles de participation pour assurer le portage d'actions ou de parts sociales, ou encore aux sociétés civiles immobilières, de plus en plus souvent propriétaires de l'immobilier d'entreprise. Au cours des dernières décennies, plusieurs textes ont permis de faire évoluer le droit des sociétés, toujours dans le sens de la simplification. Mais on doit bien constater que, parallèlement, d'autres dispositifs ont été introduits dans des lois qui n'étaient pas spécifiques aux sociétés et sont venus toucher de manière négative la vie des entreprises, en alourdissant formalisme, réglementations et contraintes diverses. Je ne suis pas sûr que sur cinq ans, dix ans ou vingt ans, la balance entre simplification et complexification soit positive, ou même simplement neutre.

En effet, depuis cette période, un certain nombre de modifications ou dispositifs proposés ont pu être partiellement ou en totalité introduits dans différents textes, en particulier la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, dite loi Macron, la loi Sapin II, la loi Pacte, ou encore les lois de finances successives. Par ailleurs, de nouvelles dispositions ont pu être introduites à l'occasion de la navette parlementaire. Sur le plan législatif, un tel processus n'est pas sérieux. En effet, en cinq ans, le contexte et l'environnement économique, technologique ou international ont changé, qui peut rendre certaines mesures obsolètes. Et encore, nous avons la chance d'avoir conservé pendant ce laps de temps les deux principaux protagonistes de cette proposition de loi

La plupart des réformes que nous engageons par voie législative reposent trop souvent sur des textes fourre-tout qui manquent généralement de ligne directrice et qui n'introduisent que très rarement des modifications en profondeur, se limitant fréquemment à des adaptations superficielles ou d'importance marginale.

une telle situation est, pour le législateur, voire pour les entreprises, un peu frustrante, car d'autres approfondissements et enrichissements du texte auraient été souhaitables et auraient permis de lui redonner une colonne vertébrale. Même si Même si certaines dispositions introduites par le Sénat n'ont pas été retenues par l'Assemblée nationale, il demeure sur l'essentiel une très large convergence entre nos deux assemblées. Je note au passage qu'a été traitée la possibilité pour des actionnaires minoritaires de demander la désignation d'un commissaire aux comptes dans des sociétés qui n'y sont plus obligatoirement assujetties. assujetties. Il est vrai que ce sujet n'avait pas été complètement apuré lors des discussions passionnées de la loi Pacte sur le seuil d'intervention des commissaires aux comptes. Je n'évoquerai pas d'autres exemples précédemment mentionnés. Mais je retiens avec satisfaction que, dans les assemblées d'actionnaires, on ne procédera pas à l'interprétation des abstentions, qui ne peuvent effectivement pas être assimilées à des votes positifs plus qu'à des votes négatifs, la neutralité étant la vocation même de l'abstention ou du vote blanc.

de cette proposition de loi Madame la présidente, madame la secrétaire d'État, mes chers collègues, la simplification de la vie des entreprises est un enjeu d'actualité fondamental pour notre économie. Il nous faut faire évoluer le code de commerce, car de nombreuses formalités inutilement lourdes et complexes pèsent en effet sur les sociétés. Viennent s'y ajouter des obligations parfois ambiguës, incohérentes, voire obsolètes. En conséquence, c'est un sentiment d'insécurité juridique qui prédomine parfois et persiste pour une partie des sociétés françaises. Et comme vous le savez, l'incertitude est l'ennemie des entreprises. À la suite du travail réalisé au sujet de la loi du 2 janvier 2014 habilitant le Gouvernement à simplifier et sécuriser la vie des entreprises, notre collègue Thani Mohamed Soilihi avait judicieusement cerné les besoins des sociétés civiles et commerciales. Les propositions à l'origine de ce texte reflètent des besoins parfaitement identifiés ; je tiens à l'en remercier. Nous sommes aujourd'hui en 2019, et je vous parle de besoins exprimés bien avant l'année 2014. Ces besoins ont-ils disparu ? Je ne le crois pas. Sont-ils devenus plus pressants ? J'en suis persuadé. Il est grand temps de répondre aux attentes des entreprises sur différents éléments qui n'ont pas été véritablement satisfaites ni par la loi Macron, ni par la loi Sapin II, ni par la récente loi Pacte, ni par les dernières lois de finances. L'environnement économique est systématiquement en mouvement. Il revient donc aux parlementaires de continuellement traquer les ajustements qui permettent de rétablir un équilibre en perpétuelle oscillation. par conséquent à saluer le travail du rapporteur, qui a su inscrire les mesures de cette proposition de loi dans la continuité des précédents textes dont il fut aussi le rapporteur. La loi du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et la loi du 10 mai 2016 ratifiant l'ordonnance du 10 septembre 2015 portant réduction du nombre minimal d'actionnaires dans les sociétés anonymes non cotées m'apparaissent comme une base solide, qu'il convient de compléter en tenant compte des avancées obtenues par les textes que j'ai préalablement mentionnés. C'est donc dans la continuité de ces avancées législatives que s'inscrit la la présente proposition de loi. En se cantonnant au droit des sociétés, les mesures qu'elle contient nous garantissent une structure cohérente. Lorsque j'analyse plus précisément le contenu de la proposition de loi telle qu'elle nous est présentée, je me réjouis que certaines dispositions adoptées sur l'initiative du Sénat aient été conservées. Et je partage avec vous, monsieur le rapporteur, quelques désaccords au sujet de certains choix de l'Assemblée nationale. Néanmoins, il faut saluer le compromis raisonnable que nos deux chambres ont pu trouver.

Nous regrettons simplement la suppression de certaines propositions qui permettaient, par exemple, d'assouplir l'échange d'informations provenant des commissaires aux comptes, ou encore d'aligner le régime applicable le régime applicable aux entités tenues d'établir des comptes combinés avec celui des entités qui sont chargées d'établir les comptes consolidés. j'estime que nous pouvons nous satisfaire des avancées, bien qu'incomplètes, de l'article 33 relatif à la simplification du régime des rachats d'actions des sociétés non cotées. Même si des améliorations restent possibles, je salue également le compromis trouvé sur l'article 23, relatif à la suppression du droit d'opposition à la dématérialisation des assemblées générales ordinaires dans les sociétés anonymes non cotées. Assouplir certaines règles de fonctionnement des sociétés ne peut être bénéfique, puisqu'il est question ici de dématérialiser la tenue des assemblées générales des sociétés anonymes, en utilisant, par exemple, les outils de visioconférence ou de télécommunication. Enfin, certaines procédures lourdes et complexes sont allégées. Je salue donc les avancées à l'article 18, qui a été plusieurs fois amendé, et dont les dispositions visent à faciliter les conditions d'octroi de cautions, d'avals ou de garanties par une société mère à ses filiales. Mes chers collègues, le groupe Union Centriste, vous l'avez compris, votera en faveur de ce texte, dont les mesures répondent aux attentes et aux besoins des entreprises. Il était absolument nécessaire de s'atteler à une clarification et à une actualisation du code de commerce. Nous ne pouvons pas attendre plus longtemps l'entrée en vigueur de ces mesures, de même que nous devrons très vite nous pencher sur les dispositions futures qui maintiendront le dynamisme de notre tissu économique. La parole

Je me réjouis que ce texte soit en discussion, près de quatre ans et demi après son dépôt au Sénat. Il était temps ! Pour le groupe Les Républicains, toutes les démarches de simplification sont bonnes à prendre, tant elles sont nécessaires. Il faut en effet desserrer les contraintes qui étouffent les entreprises pour rendre celles-ci plus compétitives, réaliser des économies budgétaires et libérer l'initiative entrepreneuriale.

Par ailleurs, selon le dernier classement d'octobre 2018 de la compétitivité économique des nations du Forum économique mondial, la France, pour l'année 2018, est à la dix-septième place sur 140, loin derrière l'Allemagne, qui occupe la troisième place.

C'est une politique économique qui place les entreprises au coeur de la croissance et qui leur donne les moyens de se développer et de créer des emplois que nous devons résolument mettre en place. C'est parce qu'elle réalise des bénéfices importants qu'une entreprise peut investir, innover, gagner des parts de marché et donc créer des emplois. Voilà pourquoi il faut continuer à réduire les charges sociales, le coût du travail et les impôts de nos entreprises. Le poids des normes et charges administratives constitue un vrai sujet. Selon une étude récente, les dirigeants de TPE-PME passeraient en moyenne deux jours par mois, soit plus d'un mois ouvré dans l'année, à effectuer des tâches de gestion juridique et administrative ! C'est une vraie perte de temps. Ces périodes devraient être consacrées à des missions plus rentables et génératrices de valeur ajoutée.

La France doit redevenir attractive économiquement. Pour ce faire, il faut simplifier les contraintes administratives qui pèsent sur les chefs d'entreprise et accompagner ces derniers. Soyons aussi attentifs à ne pas modifier constamment la politique fiscale et juridique des entreprises : elles ont également besoin de stabilité. C'est l'objet de ce texte, texte, qui vise à simplifier les dispositions du code de commerce et du code civil devenues trop complexes, désuètes ou lacunaires, tout en assurant aux acteurs économiques une certaine stabilité de leurs règles de droit et en préservant la protection des intérêts des tiers- salariés, actionnaires, clients et fournisseurs. Du fait de l'importance du délai entre son dépôt et son examen, le texte a subi des modifications et des suppressions de dispositions et d'articles prévus et adoptés dans le cadre d'autres lois. Ainsi, de nombreuses mesures ont été reprises dans la loi du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques et dans la loi du 10 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

Cette proposition de loi s'inscrit dans le processus permanent de simplification du droit des entreprises engagé depuis de nombreuses années. Elle s'appuie notamment sur les travaux du Conseil de la simplification pour les entreprises, qui a été créé par décret au mois de janvier 2014 pour une durée de trois ans qui était chargé de proposer au Gouvernement les orientations stratégiques de la politique de simplification à l'égard des entreprises. Elle est étroitement liée à la loi Pacte, dans la mesure où cette dernière a pour ambition de donner aux entreprises les moyens d'innover, de se transformer, de grandir et de créer des emplois. Les grands sujets abordés par le texte comprennent en particulier le régime des fonds de commerce, sur lequel aucune disposition ne demeure en discussion, une modernisation des dispositions du code civil et du code de commerce relatives aux sociétés civiles et sociétés commerciales, notamment une simplification des obligations formelles imposées aux sociétés. l'ajout de dispositions plus spécifiques aux cas de tutelle des responsables de société. Cette mesure, tout particulièrement attendue par les notaires, est un élément assez important du texte, dont l'objectif est de remédier aux situations de blocage dans certaines petites entreprises qui peuvent naître de la mise sous tutelle du gérant. Jusqu'à présent, la procédure prévue dans le code de commerce ne permet le remplacement de ce dernier qu'en cas de décès. Le texte propose aussi une clarification de certaines dispositions concernant les commissaires aux comptes. Parmi les mesures adoptées par l'Assemblée nationale, j'aimerais relever un élément qui me semble intéressant et assez parlant : la facilitation de la dématérialisation des assemblées générales ordinaires des actionnaires des sociétés Toutes ces dispositions vont dans le bon sens. La simplification et l'actualisation d'un texte de loi sont souvent les bienvenues, notamment lorsqu'elles ont trait à des mesures lourdes, ambiguës et contraignantes pour les personnalités physiques ou morales. Ce texte touche à des dispositions du droit des sociétés qui nécessitaient d'être actualisées, afin de fluidifier la vie des entreprises et les relations économiques. Tout cela semble parfaitement justifié. C'est pourquoi le groupe Les Républicains votera le texte en l'état. La discussion

au bout de quelques mois avec cinquante salariés sans que l'on puisse assurer la coordination entre les moyens de la société, les comptes courants et, éventuellement, le paiement de charges

le Sénat que la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi d'orientation des mobilités n'est pas parvenue à l'adoption d'un texte commun.